dans l'analyse politique du scrutin. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

est tenu de solliciter l'avis du préfet. Mais cet article ne prévoit cette procédure que pour les permis de construire et les déclarations de travaux, sans qu'il soit fait mention du certificat d'urbanisme opérationnel.

Mais l'apparition du certificat d'urbanisme opérationnel les a rapprochés effectivement d'un permis ou d'une décision de non-opposition. Sur cet amendement, je sollicite l'avis du Gouvernement.

le règlement national d'urbanisme s'applique à nouveau sur le territoire communal s'il n'existe pas de document d'urbanisme antérieur. Les demandes d'autorisation d'urbanisme sont alors soumises à l'avis conforme du préfet. Le certificat d'urbanisme, lui, n'y est pas soumis ; il doit simplement indiquer que cet avis devra être recueilli au stade de la demande de permis.

il n'est porté qu'une appréciation très relative sur la faisabilité du projet- la localisation approximative, par exemple. Même si le préfet intervient à ce moment, rien ne garantit la délivrance ultérieure de l'autorisation. Les services préfectoraux doivent se concentrer de manière privilégiée sur ce qui présente de véritables enjeux pour l'État. Systématiser l'avis conforme du préfet, c'est-à-dire son accord

effet que, en amont des projets, un dialogue est noué entre le porteur de projet, l'État- sous l'autorité du préfet -et la collectivité. Cela permet effectivement

ville. L'amendement que nous avions déposé n'a pas été voté, les ministres nous ayant dit, ce dont nous prenons acte, que tous les outils existent aujourd'hui pour permettre que ces espaces évoluent dans le bon sens.

l'avis du Gouvernement ? Je n'ai jamais été très favorable aux rapports et à leur multiplication. Je ne changerai pas d'avis, même si j'ai changé de fonctions.

et des possibilités d'amélioration du cadre de vie, du paysage architectural, des entrées de ville, le Parlement a tous les moyens d'oeuvrer utilement. Nous ferons le meilleur usage

mes chers collègues, nous abordons, avec cet article et les suivants, la problématique de l'urbanisme en milieu rural. Sans reprendre les débats que nous avons eus ici hier après-midi et hier soir, je veux simplement rappeler que, pour notre groupe, l'objectif n'est pas d'interdire la construction en zone rurale ; en revanche, nous ne voulons pas permettre une dérégulation et une déréglementation totales qui fragiliseraient la construction pour les décennies à venir dans nos territoires ruraux. Nous pensons, et nous l'avons toujours dit ici, que c'est non pas de déréglementation, mais bien de moyens humains et financiers pour maintenir un niveau acceptable de services publics dont ont besoin les territoires ruraux dans notre pays. Les problématiques de logement ne peuvent s'appréhender séparément des enjeux de mobilité, de déplacement, de développement économique,

entre les territoires, voulant rompre justement avec cette mise en concurrence des territoires et des hommes et tordre le cou finalement à l'hypermétropolisation qui s'installe dans notre pays, année après année. C'est bien de cela qu'ont besoin nos territoires, des territoires parfois enclavés. Ils ont besoin d'un effort de la puissance publique pour garantir l'égalité républicaine à toutes et à tous, quelles que soient leurs conditions sociales, mais aussi quelles que soient leurs conditions territoriales. Pour notre part, nous nous opposons à un usage dispendieux des terres agricoles et naturelles. Nous ne sommes pas des ayatollahs de tel ou tel principe ou de telle ou telle posture dogmatique, mais nous considérons que le foncier est un bien rare et précieux qu'il convient d'utiliser au plus juste et qu'il ne faut pas produire des politiques d'artificialisation des sols aux conséquences Nous avons débattu hier des territoires à aménager. Bien évidemment, il faut permettre aux territoires ruraux de se développer et de construire, limiter également l'invasion par la forêt, nuisible dans un certain nombre de nos villages, mais aussi réglementer pour empêcher de faire tout et n'importe quoi et de détruire la qualité de

Les textes permettent actuellement de réaliser des extensions ou annexes aux seuls bâtiments d'habitation. Par ailleurs, la commission a prévu que ces nouvelles possibilités de constructions s'appliqueraient également aux communes n'étant couvertes par aucun document d'urbanisme. De fait, ces constructions nouvelles pourraient n'être encadrées par aucun document d'urbanisme et l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, la CDPENAF, serait supprimé. Ces dispositions marquent un recul important pour la protection du foncier agricole, alors que tous s'accordent à dire que ces zones agricoles sont des zones pour lesquelles la constructibilité doit rester très limitée. Est-il nécessaire de rappeler que c'est dans ce monde rural que la surface imperméabilisée par habitant est la plus forte Il semble qu'aujourd'hui la nécessité pour les communes d'élaborer un projet de territoire économe en matière de consommation foncière ne fait plus débat. C'est la raison pour laquelle nous devons encourager les communes à se doter d'un document d'urbanisme qui permettra aux maires d'élaborer leurs projets de développement et de choisir ainsi leur avenir, plutôt que de le subir. Cet article 12 est donc un très mauvais signal à la fois pour l'aménagement et la planification, mais également pour l'activité des territoires. C'est pourquoi nous en demandons la suppression. Quel est

adoptée par la commission, est de nature à faciliter la réalisation de travaux de faible ampleur, tels que la construction d'annexes. Elle garantit que les constructions édifiées ne porteront pas atteinte aux paysages et aux espaces naturels,

12 corrigeait une erreur qui avait vicié la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture Nous avions la volonté de rétablir la possibilité d'autoriser les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles dans les secteurs non constructibles. La commission des affaires économiques

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

Cet amendement vise à simplifier le fonctionnement d'installations directement liées à l'activité agricole et à en diminuer l'impact environnemental. Les stockages, qu'ils soient liés à des besoins locaux ou autres, nécessitent de se trouver au coeur des productions de cultures afin de limiter les coûts temps-distances des exploitants agricoles et le nombre de rotations des engins agricoles, encombrants, lents et lourds, qui est nettement plus important que celui des poids lourds distribuant les productions concentrées. Les rotations des engins agricoles peuvent atteindre des dizaines de véhicules sur les périodes de récoltes et ainsi provoquer des gênes sur des voies de faibles largeurs, des ralentissements importants et abîmer nos routes départementales ou communales. De plus, le nombre de rotations diminuant, l'impact carbone en sera d'autant plus réduit. Enfin, sortir les silos et autres éléments de stockage agricoles des zones d'activité économique permet d'éviter les contraintes liées à leur affectation en installation classée. Dans les zones artisanales, équipées et donc plus onéreuses, des distances de sécurité sur des rayons importants impliquent l'absence de toute construction et grèvent ainsi des surfaces importantes, qui auraient pu trouver une autre vocation. C'est pourquoi le présent amendement

Cet amendement vise à autoriser les silos commerciaux dans les zones inconstructibles des cartes communales, alors que ces silos ne sont pas autorisés

permet à la carte communale de délimiter des secteurs réservés à l'implantation d'activités, « notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». La délimitation

liste les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font seulement l'objet d'une déclaration préalable. Ainsi, dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d'urbanisme, la construction d'extensions inférieures ou égales à 40 mètres carrés de surface de plancher ne requiert qu'une déclaration préalable, alors que dans les autres zones, dès 20 mètres carrés, il est nécessaire de déposer une demande de permis de construire. Toutefois, si l'extension, comprise entre 20 et 40 mètres carrés, aboutit à ce que l'ensemble de la construction excède le seuil de recours obligatoire à un architecte, un permis de construire avec l'intervention d'un architecte est requis. Or le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 a abaissé à 150 mètres carrés, au lieu de 170 mètres carrés, le seuil de recours obligatoire à un architecte pour les particuliers. L'abaissement de ce seuil a considérablement augmenté le nombre de cas où des extensions inférieures à 40 mètres carrés sont soumises à un permis de construire signé par un architecte, alors qu'auparavant une simple déclaration préalable suffisait. Ce surcoût lié à l'intervention de l'architecte remet bien souvent en cause la réalisation des travaux. Les entreprises intervenant sur le secteur des travaux de rénovation/extension sont extrêmement inquiètes pour la pérennité de leur activité. C'est pourquoi il serait judicieux que, dans les communes couvertes par un PLU, les travaux d'extension d'une construction existante créant jusqu'à 40 mètres carrés de surface de plancher soient systématiquement soumis à déclaration préalable. C'est une question de bon sens à partir du moment où le Gouvernement a modifié la surface prise en compte.

il faut un permis de construire, avec intervention d'un architecte, qui reste nécessaire à partir d'une extension de 20 mètres carrés. De plus, il faut être conscient que la règle actuelle est indispensable pour limiter les risques de fraudes

des parcelles de terrains situées en plein centre de zones précédemment urbanisées, communément appelées « dents creuses ». Pourtant, ces espaces inoccupés bénéficient dans la plupart des cas de réseaux et de voiries réalisés par les collectivités territoriales. Ils sont malheureusement voués à la friche et à l'abandon, car manifestement inappropriés à un usage agricole. Ces espaces peuvent être très facilement recensés à l'échelle de chaque commune lors de l'élaboration des documents d'urbanisme- schéma de cohérence PLU, PLUI. Aujourd'hui, la loi nous prescrit de densifier les zones urbanisées et de préserver l'espace agricole. C'est bien dans cet esprit que j'ai déposé un amendement qui a été adopté par la commission et donc pris en compte dans l'article concerné. Une telle disposition offrirait plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permettrait d'optimiser un potentiel foncier intéressant qui peut avantageusement fixer, voire accueillir, de nouvelles populations dans des zones menacées de désertification. Elle permettrait aussi de limiter, sans les interdire, les extensions dans le périmètre rapproché des bourgs ou des centres-villes et serait donc un frein à la réduction foncière de l'espace agricole. N'oublions pas que, dans certaines situations, plus le périmètre d'imperméabilisation d'un bourg et d'une agglomération est important et dense, plus les risques d'inondation sont élevés. Enfin, et les élus locaux que nous sommes ou que nous avons été y sont sensibles, elle permettrait de ralentir, à défaut d'y mettre un terme, les multiples contentieux auxquels ont à faire face de très nombreux maires de France, certains, de guerre lasse, finissant par jeter l'éponge. Monsieur le ministre, il me semble important d'indiquer qu'il faut lever l'instabilité du caractère exceptionnel, qui donne la part belle à l'administration ou au juge administratif. Cet amendement est un ajustement de la loi après quatre années d'application et deux rapports parlementaires pointant cette situation. C'est le problème que j'évoquais dans mon intervention du 26 octobre 2017. Aussi, je me permets de vous rappeler deux phrases de votre réponse, Monsieur le sénateur, vous avez raison, il ne faut pas toujours se cacher derrière des arguments. L'ingénieur agronome que je suis n'ignore rien de l'artificialisation des terres agricoles. Il n'empêche que l'artificialisation des zones agricoles ne se fait pas au centre d'un hameau, comme vous l'avez dit. Les dents creuses aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, la loi ALUR les permet déjà, dès lors qu'il s'agit d'un bâti. La question qui se pose est : pouvons-nous élargir le dispositif au foncier et ne pas le limiter uniquement au bâti ?

ou forestière, l'article 19 de la loi Grenelle I a consacré la possibilité pour le plan local d'urbanisme de délimiter des secteurs de taille et de capacité limitées. Il s'agit donc d'une dérogation au principe de l'urbanisation limitée et consécutive. Toutefois, la loi ALUR a apporté une restriction significative au dispositif des STECAL en indiquant qu'il s'agit d'une modalité acceptée à titre exceptionnel. Ainsi, il ne peut y avoir, selon les services de l'État, plus de deux STECAL sur le périmètre d'une intercommunalité. Je suis bien d'accord, le regroupement intercommunal forcé, voulu et voté par certains, à une échelle très importante, n'est pas sans poser des questions aujourd'hui. Cependant, avec l'amendement qui a été adopté par la commission des affaires économiques du Sénat, il s'agit à nos yeux, sous couvert de sécurisation juridique, de rouvrir grand la porte à la multiplication de ces STECAL. Cela revient en réalité à supprimer cette modalité d'exceptionnalité. On est donc loin,

témoigne de la volonté de sécuriser ces réalisations, nous pensons au contraire que cela crée une insécurité juridique manifeste. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article 12 A, tel que rédigé à l'issue des travaux de la commission des affaires économiques.

Notre amendement vise à supprimer la définition du caractère exceptionnel des STECAL introduite par la commission des affaires économiques. Mon argumentation est la même que celle qui a été développée par la sénatrice Cécile Cukierman, car l'état actuel du droit n'apporte pas de précision sur la notion de caractère exceptionnel du secteur, qui peut cependant être apprécié dans le PLU en fonction des spécificités de chaque territoire et complété lors de son examen obligatoire par la

Duran, pour présenter l'amendement n° 550. Actuellement, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole sont permises. C'est l'article L. 311-1 du code rural qui définit la notion d'activité agricole, à savoir les activités exercées exercées dans le prolongement de l'exploitation agricole, telle la vente des produits de la ferme, ou ayant pour support l'exploitation- gîtes ruraux, agritourisme, hébergement touristique, etc. La commission des affaires économiques a voulu aller plus loin en autorisant les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou encore en vue d'une activité d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, notamment pour l'hébergement et la restauration. Ces constructions seraient rendues possibles y compris en RNU- règlement national d'urbanisme -donc sans encadrement par un document d'urbanisme. Les évolutions récentes ont permis de trouver un équilibre entre l'impératif d'une gestion économe de l'espace agricole, le maintien

de développer nos territoires, que plus personne ne peut construire nulle part, que tous les agriculteurs sont bloqués dans leur développement. Telle serait la réalité de la France, d'un pays qui s'effondre. Et, de leur côté, les autres regardent le monde

peuvent déjà être autorisées, sur délibération motivée du conseil municipal, dans les communes qui sont en règlement national d'urbanisme, ainsi qu'à l'intérieur des STECAL pour les communes qui sont couvertes par un PLU. Aujourd'hui, l'autorisation

Cet article vise à rationaliser la procédure de consultation de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, la CDPENAF, pour ce qui concerne les dérogations à l'interdiction de construire hors des parties urbanisées des communes. par l'Assemblée nationale, il visait initialement à regrouper deux procédures qui nécessitaient les mêmes autorisations, lorsqu'une commune n'était couverte ni par un PLU ni par un SCOT.

l'avis conforme de la CDPENAF. Il s'agit, premièrement, du changement de destination d'un bâtiment en zone agricole d'une commune disposant d'un PLU ; et, deuxièmement, des constructions d'intérêt communal hors zone urbanisée d'une commune soumise au RNU.

nous estimons que, lorsque ces dérogations ont pour conséquence de réduire les surfaces à vocation agricole des zones non urbanisées, la commission départementale a un rôle fondamental à jouer. En passant d'un avis conforme à un avis simple, on permet clairement aux maires le moins excessif ! ... ce qui n'est pas toujours souhaitable. Nous ne souhaitons pas un développement urbain à outrance. Nous restons attachés au principe d'une urbanisation limitée dans ces zones,

l'avis conforme, l'on sécurise également le maire dans son rôle, dans sa capacité à décider en lien avec les services de l'État, et l'on évite les dérives que l'on a pu constater dans l'ensemble des territoires.

hors des parties urbanisées des communes non couvertes par un SCOT, des constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et de leur extension mesurée, ainsi que des constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, visées au 4° de l'article

ce n'est pas simple tous les jours. Il faut prendre en compte des réalités, des rapports de force,

qui sont tout à fait conscients de la nécessité de protéger la nature. N'y a-t-il pas dans notre pays deux poids, deux mesures ? D'un côté, de grands ensembles n'en finissent pas de prolonger, en région parisienne ou ailleurs, l'espace urbain

par le fait que, dans le domaine rural, tout est interdit, ou presque. Comme en toute chose, il faut raison garder : on ne peut pas tout autoriser d'un côté, rien de l'autre ! Sans activité économique, les territoires ruraux finiront par se vider de leurs habitants. L'article 12 rationalise la procédure de consultation de la CDPENAF et répare une injustice dont souffrent les communes rurales et les hameaux où il y a des dents creuses.

ne revêtir qu'un caractère exceptionnel, afin d'éviter l'aggravation du mitage et de la perte de vocation des espaces naturels et agricoles, par nature inconstructibles. En outre, de tels projets peuvent entraîner une perte importante de surfaces agricoles ou naturelles. Or, aujourd'hui, le code de l'urbanisme offre la possibilité d'autoriser de telles constructions les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, les STECAL, autorisés par une procédure de révision du PLU. devant être précisément mesuré et débattu avec la population et les élus, une procédure de modification simplifiée hors STECAL paraît contraire à l'objectif de protection de ces espaces. C'est pourquoi nous souhaitons le retour au dispositif initial. Je mets

dériver la jurisprudence, qui aujourd'hui rend les choses impossibles. Les maires sont dans une insécurité juridique totale, et les communes littorales sont bloquées sur un certain nombre de sujets, y compris les professionnels.

la modification législative des excès de la jurisprudence sur la loi Littoral

certes précaire, entre la préservation nécessaire de nos littoraux et la prise en compte de la démographie croissante à laquelle doit faire face notre pays. À cet effet, cette loi se fondait sur deux principes : un développement urbain uniquement dans la continuité des villes et villages existants et la protection, pour des raisons environnementales et esthétiques, des littoraux sur un espace

L'intention est bien sûr louable : nous avons, certes, besoin de plus de services publics et de logements plus nombreux, notamment pour les plus précaires. Toutefois, cette solution comporte un écueil de taille : elle est la porte ouverte à toutes les dérives. En effet, si une dérogation était consentie pour le service public et le logement social, qu'est-ce qui empêcherait, plus tard, la prolifération sur les littoraux de complexes hôteliers ou de locaux relevant du secteur privé ? Alors même que la loi ALUR permet déjà un certain nombre de dérogations, fermement encadrées, afin de densifier et d'améliorer l'offre de logements, l'exécutif, probablement au service de lobbies de l'immobilier,

a dit voilà plus d'un an Emmanuel Macron, exhortant les chefs d'État du monde à respecter leurs engagements internationaux en matière environnementale. Cela ne concernait de toute évidence pas la préservation de nos littoraux ...

qu'il importe, à mon sens, de tenir compte de la réalité de ce que connaissent les élus qui vivent les questions liées à la loi Littoral. Je n'aimerais pas que ceux d'entre nous qui ne connaissent pas ni ne pratiquent la loi Littoral viennent faire la leçon à ceux qui connaissent les problèmes au jour le jour.

Littoral : « Mais vous n'êtes pas non plus tombés dans le conservatisme qui fait que, tout en protégeant légitimement la côte, le littoral, plus aucun projet ne serait possible. Je sais, nous l'avons vu hier encore, que certains élus ont vécu avec cruauté- nous en parlions ce matin -les projets qui ont pu être bloqués, parce que, progressivement, nous avons construit ce qui est sans doute une vision excessive de la fameuse loi Littoral. Mais tout cela, c'est quoi ? C'est le fruit d'une vision qu'on n'arrive plus à expliquer avec bon sens. On veut protéger le littoral, et nous allons continuer à le faire. La loi Littoral est une bonne loi et sera préservée, mais elle a des aberrations. Quand un acteur économique ou touristique est là de tout temps et qu'il lui faut revoir ses structures, les étendre un peu dans le cadre des documents d'urbanisme pris en vertu de la loi, donc dans le respect de ladite loi, il faut qu'on puisse trouver les bons aménagements. Lorsqu'on demande à une station d'épuration ou un centre nautique d'être réhabilité et qu'on lui dit : à cause de la loi Littoral, ce ne sera plus possible, on ne peut pas expliquer légitimement, face aux jeunes qu'on ouvre à la mer et au goût de la mer, qu'on va encourager ce goût en fermant le centre nautique. Il faut, là aussi, un peu de pragmatisme et de bon sens. Je crois que vos élus en ont et je pense que les avancées commencées à l'Assemblée nationale seront poursuivies au Sénat pour permettre de traiter ce sujet. » « Et l'autre sujet que, je dois dire, j'ai découvert il y a près d'un an chez vos voisins du Morbihan- Jacques Le Nay était là tout à l'heure -, c'est ce fameux sujet des dents creuses, une spécialité pas tout à fait uniquement bretonne, ... Également corse ! ... mais très bretonne, qui là aussi est un peu une aberration de la loi Littoral

Les dispositions introduites sont des mesures d'équilibre qui ne remettent aucunement en cause les fondements de la loi Littoral, contrairement à ce qu'on a prétendu, mais visent à définir des règles d'urbanisation claires afin de mettre fin aux lourdes difficultés rencontrées par les propriétaires des terrains concernés, ainsi que par les maires, qui font face à de nombreux contentieux en la matière. en la matière. Le code de l'urbanisme prévoit jusqu'à présent que, dans les communes littorales, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

La notion de hameaux n'est en effet pas satisfaisante, car des dents creuses existent également dans des secteurs qui ne peuvent être qualifiés d'agglomérations ni de villages existants, mais qui sont trop importants pour être qualifiés de hameaux. En outre, avec l'introduction de cet article 12 , c'est le SCOT qui aura la responsabilité de définir les zones où pourront être comblées les dents creuses. Seuls des logements et équipements de service public pourraient être construits ou installés dans ces dents creuses. L'autorisation serait refusée si ces constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou au paysage. La possibilité de densifier les formes urbaines intermédiaires entre le village et l'urbanisation diffuse ne s'appliquera ni dans la bande des 100 mètres ni dans les espaces proches du rivage.

de révision de ces documents longue- plusieurs années -et coûteuse- plusieurs centaines de milliers d'euros -pour les collectivités territoriales, en prévoyant la possibilité de recourir, jusqu'au 31 décembre 2021, aux procédures de modification simplifiée prévues par le code de l'urbanisme. De même, la durée du dispositif transitoire institué dans cet article a été allongée jusqu'au 31 décembre 2021, afin de permettre aux préfets de débloquer la situation locale. Nous soutenons donc l'ensemble de ces dispositions et souhaitons un large soutien à l'article 12 au sein de notre hémicycle ! Très bien

de considérer que nous sommes collectivement capables de défendre un bien commun, là où beaucoup d'autres ont échoué, du fait de la pression des intérêts privés et de la perméabilité des élus locaux à ces intérêts. Je ne ferai pas la liste complète et je ne serai pas trop donneur de leçons pour les pays alentour. Ils ont, en tout cas, détruit leur bien commun. La loi Littoral, c'est ainsi la force de la société française. C'est pourquoi, comme dirait le président Larcher pour la Constitution, il ne faut y toucher que d'une main tremblante.

État et associations de protection de l'environnement et du patrimoine peuvent se mettre d'accord sur une dérogation pour laquelle il y a consensus, on aura toujours des difficultés avec la loi Littoral.

de la loi Littoral n'interdit la construction dans les dents creuses : c'est une construction des jugements de tribunal administratif, et, d'ailleurs, il y a eu dans la jurisprudence de ces tribunaux de grandes différences d'appréciation. Il s'agit d'une manière limitée et en protégeant ce bien commun, de faire en sorte que, sans être sur le rivage, sans avoir vue sur la mer et à l'intérieur de hameaux déjà construits, sur des terrains qui sont encadrés par deux constructions existantes, on puisse désormais construire. Dans le département de la Manche, nous avons le deuxième plus long littoral de France métropolitaine. Nous cherchons bien sûr à le protéger, car c'est notre richesse, mais nous ne pouvons absolument pas continuer à accepter que des retraités qui ont acheté un terrain constructible voilà vingt ans, alors que la loi Littoral était déjà applicable, ne puissent pas

à ces difficultés qui n'ont que trop duré, pour rendre la justice en faveur des propriétaires de ces petits terrains : ils devront pouvoir construire demain, sur autorisation du préfet et avec des documents d'urbanisme qui le leur permettront

L'article 12 prévoit plusieurs évolutions, dont le remplacement de la notion de « hameaux nouveaux intégrés à l'environnement », appréciée de manière extrêmement limitative par la jurisprudence, par celle de « secteurs déjà urbanisés », qui s'oppose à l'urbanisation diffuse. Pour notre part, nous estimons que des évolutions sont envisageables et nous en avons proposé. En particulier, nous considérons qu'il vaut mieux densifier là où il existe déjà des éléments bâtis avec un caractère structuré et regroupé plutôt que d'empiéter sur des zones non urbanisées. Dans ce cadre, la disparition de la notion de « hameaux nouveaux » nous convient. Pour autant, comme nous l'avons déjà dit, nous aurions aimé que soit mené un travail de définition sur les notions qui conditionnent la possibilité de construction dans ces zones. Nous souhaitons ainsi que soient définies les notions d'agglomération, de village, mais également de zone déjà urbanisée, ce qui permettra de prendre en compte les hameaux déjà construits où se situent les dents creuses. La jurisprudence concernant la loi Montagne est plus claire. Nous savons, par exemple en Isère, qu'un groupement est constitué à partir de quatre maisons distantes de moins de cinquante mètres, et que dans ce cadre, et uniquement dans ce cas, il est possible de densifier. La définition actée dans le présent article issue des travaux de la commission est trop large. Il s'agit de secteurs « qui se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipement ou de lieux collectifs ». Rien donc sur le caractère regroupé des habitations. Une telle définition, qui donne la responsabilité aux SCOT de localiser ces zones, semble ouvrir la voie à une urbanisation trop large, atomisant ainsi la loi Littoral. Nous proposons donc la suppression de cet article.

dans bien des endroits, la tentation de construire tout près du bord de mer plutôt que de revaloriser de petits villages proches dans les terres n'est pas une bonne idée pour le développement de notre pays.

qu'il ne s'agit ni d'affaiblir la loi Littoral ni d'un passage en force comme on peut l'entendre, mais qu'il s'agit simplement de trouver des solutions précises et encadrées à des problèmes précis

encadrée mais territorialisée les documents locaux d'urbanisme. Cela va justement dans le sens de la proposition de loi de Michel Vaspart. Les constructions limitées et n'étendant pas l'urbanisation seront permises dans les secteurs qui sont déjà urbanisés avec avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Arrêtons de faire des procès

La position du Gouvernement a été clairement exprimée à l'Assemblée nationale. Nous sommes très attachés à la loi Littoral,

Nicolas Hulot et Jacques Mézard saluent le travail du Parlement pour préserver la loi Littoral et prendre en compte les réalités locales ». Mais bien sûr !

ce serait contradictoire avec la position du Gouvernement dans le débat qui s'est tenu précédemment à l'Assemblée nationale. En revanche, nous ne sommes pas d'accord avec toutes les évolutions qui sont proposées par la commission sénatoriale. sénatoriale. Nous aurons donc à exprimer notre position au cas par cas, mais globalement, telle est la position du Gouvernement : ne pas être bloqué, et nous l'avons montré, sur la question des dents creuses et trouver des solutions

-conduit à de grandes difficultés de développement pour ces territoires relevant à la fois de la loi Montagne et de la loi Littoral. Aux termes de la loi Littoral, les seules possibilités d'extension doivent se faire soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. La définition d'une agglomération, d'un village ou d'un hameau est explicitée dans l'instruction du 7 décembre 2015. Or dans ces territoires spécifiques, même ce qui existe est contraint puisqu'on ne permet pas à certaines urbanisations de s'étendre.

De plus, la constructibilité en continuité n'est pas une garantie de protection des paysages et de l'environnement. La seule possibilité qui nous était offerte pour déroger à la constructibilité en continuité était la création d'un hameau nouveau intégré à l'environnement. Supprimer la possibilité de créer un tel hameau est la garantie certaine de figer un territoire, sur le plan tant résidentiel qu'économique, et plus précisément touristique, qui est un enjeu majeur des territoires de montagne. Conserver la possibilité de créer un hameau nouveau, c'est garder une chance d'évolution et de développement face à une réglementation déjà très contraignante, afin de trouver un équilibre dans le développement des territoires de montagne.

l'avis de la commission sur ces deux amendements ? Ma chère collègue, le projet de loi remplace la notion de hameau aux contours jurisprudentiels flous par la notion de secteur déjà urbanisé dont les contours seront définis par les documents locaux d'urbanisme de manière territorialisée.

En l'état actuel du droit, l'extension de l'urbanisation se réalise sur le littoral soit en continuité de village ou d'agglomération, c'est-à-dire en continuité de secteurs présentant un nombre et une densité significative de constructions, soit dans un hameau nouveau intégré à l'environnement. Or il n'existe pas

et non rétroactive, si bien que les projets qui ont déjà fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme resteront autorisés. L'objectif visé par votre amendement est donc intégralement satisfait.

par leur densité et leur caractère structuré. La commission des affaires économiques a complété l'identification de ces secteurs par les notions de densité de l'urbanisation, de continuité, de structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès Le texte adopté précise que cette liste n'est pas exclusive. Toutefois, contrairement à l'effet recherché de sécurité juridique, cette liste nous paraît être source de difficultés d'interprétation. Le présent amendement vise donc à supprimer cet ajout.

mais qui ne sont pas assimilables à un village. Dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, cet article prévoyait d'inscrire au niveau législatif deux critères minimaux- densité et structuration -pour définir les secteurs intermédiaires, et de renvoyer au SCOT le soin de préciser

mais aussi à freiner la saturation touristique de la Côte d'Azur et à accueillir de nouvelles populations. Cette initiative est toujours citée comme exemple d'aménagement du territoire réussi, puisqu'elle a permis la mise en valeur efficace d'espaces naturels peu attractifs et a rendu la mer accessible aux bénéficiaires d'un tourisme de masse planifié, au plus grand profit des touristes eux-mêmes et des activités économiques qu'ils ont contribué à développer. L'érosion et le recul du trait de côte rendent nécessaire l'actualisation des emplacements des aménagements réalisés en repositionnant ceux-ci dans des espaces correspondant à leur vocation, c'est-à-dire des secteurs déjà urbanisés

la loi Littoral, afin de permettre la relocalisation dans les espaces proches du rivage d'activités et de biens des littoraux languedociens touchés par le recul du trait de côte. Or, en l'état

qui associe espaces rétrolittoraux et interface terre-mer. Il serait donc tout à fait contradictoire que la gestion du recul du trait de côte puisse systématiquement échapper au principe d'aménagement applicable sur le littoral

de se substituer au SCOT pour déterminer les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés, dans lesquels les constructions et installations peuvent être autorisées dans les secteurs littoraux,

l'article 12 exclut la densification des secteurs déjà urbanisés dans la bande des cent mètres et dans les espaces proches du rivage. S'il n'est évidemment pas question de remettre en cause ce dispositif, deux deux problèmes demeurent : tout d'abord, celui des îles et presqu'îles, dont le territoire est intégralement compris dans les espaces proches du rivage ; le second concerne les stations balnéaires qui se sont développées avant la loi de 1986, et les lacs de montagne, que mon collègue Jean-Pierre Vial

Actuellement, si celles-ci doivent être liées à des activités agricoles ou forestières, incompatibles avec le voisinage de zones habitées, les conditions prévues sont cumulatives : ces dérogations ne peuvent pas porter atteinte à l'environnement ou aux paysages, ne peuvent être autorisées dans les espaces proches du rivage et doivent recueillir l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'article adopté par l'Assemblée nationale permet aux constructions liées aux activités agricoles ou forestières de faire l'objet de dérogations à l'inconstructibilité de zones, qui ne se situent pas dans des espaces urbanisés, même lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec le voisinage de zones habitées. On se demande pourquoi il serait nécessaire de pratiquer le mitage et l'étalement urbains pour des activités qui peuvent être poursuivies en zone urbanisée. Nous proposons donc la suppression de cet article. La

pour valoriser les zones agricoles selon leur plein potentiel. Elle impose des restrictions disproportionnées aux exploitants de cultures marines. Un assouplissement des critères, tel que le propose la commission, qui permettrait des constructions en zone non urbanisée,

12 , qui permet l'implantation, en discontinuité de l'urbanisation, des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières qui ne sont pas incompatibles avec le voisinage des zones habitées, en dehors des espaces proches du rivage, et avec

débloquer des situations qui posaient problème à nombre de collectivités locales, de communes du littoral, mais sans aller jusqu'à la remise en cause

et nombre d'amendements témoignent des inquiétudes et des questions que cette loi peut soulever. Comme l'a rappelé M. le ministre, le projet de loi initial du Gouvernement ne prévoyait aucune disposition sur la loi Littoral, qui, je le rappelle, concerne quand même 1 212 communes, 975 communes situées aux abords de la mer ou de l'océan, et 237 autres communes, que l'on oublie peut-être un peu, riveraines d'un lac, d'un estuaire ou d'un delta. Face aux débordements de l'Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé un compromis pour répondre à la question particulière des dents creuses. Le SCOT définira les zones où les dents creuses pourront être comblées. Seuls des logements et des équipements de service public pourront y être construits, mais l'autorisation sera refusée en cas d'atteinte à l'environnement et au paysage. Le Sénat a ensuite introduit une procédure de modification simplifiée du SCOT

avancées constituent une remise en cause des dispositifs fondamentaux de la loi Littoral. Or nous savons- cela a été rappelé -que cette loi est indispensable à la préservation des milieux naturels, qu'elle constitue la seule possibilité de prévenir les risques et de protéger les biens

Le travail en commission a permis d'autoriser les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines en dehors des espaces proches du rivage. Cette autorisation est très encadrée et tout changement de destination de ces constructions est interdit.

de valorisation de cultures marines, des activités qui sont souvent attachées à de petits locaux d'exploitation : ateliers conchylicoles accueillant du public, points de vente réduits de produits de la mer,

les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines, et à leur valorisation

Vaspart, je n'aurai ni la cruauté ni le temps de reprendre les déclarations et travaux des uns et des autres et de mettre en avant, avec délectation ou colère, les évolutions et changements de position,

Je vois difficilement comment on peut maintenir dans la loi cette terminologie, dont,, je perçois bien les effets et les dangers.

! C'était l'exception qui confirme la règle ! J'ai toujours été hostile à toute remise en cause de la loi Littoral ; cette affaire était momentanément passée hors de mes écrans radars.

le dire, vous a permis de marquer un point : effectivement, c'est bien vous qui représentez l'exécutif et le Président de la République, qui n'est pas responsable devant le Parlement, ne peut représenter l'exécutif devant lui. Nous sommes d'accord Nous sommes d'accord avec cette interprétation, qui émane, d'ailleurs, d'un ancien collègue parlementaire particulièrement chevronné et respecté, singulièrement au Sénat.

est-ce une interprétation un peu naïve. Mais, pour moi, quand le Président de la République s'exprime devant les députés et sénateurs d'un département, devant le maire de Saint-Brieuc, devant le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, devant le président du groupe La République En Marche de l'Assemblée nationale- le principal parti de la majorité présidentielle -et qu'il annonce sa volonté de régler ce qu'il avait qualifié, un peu moins d'un an plus tôt, d'aberration- il visait non pas la loi Littoral, mais son application -, cela devrait valoir instruction aux membres du Gouvernement, et ce même si seuls les ministres peuvent s'exprimer au nom de l'exécutif devant nous ! Il y a là, je crois, un problème dans le fonctionnement de l'État.

au fonctionnement de ces cultures marines et, bien sûr, à la valorisation des produits qui en ressortiront me paraît relever de la logique et du bon sens !

ces cultures, mais développons-les en mer ! Pour revenir à l'amendement du Gouvernement- très brièvement, puisque tout a été dit -, il serait extrêmement dangereux

qui a une telle affection pour le régime de la V République qu'il ne peut s'empêcher de la réaffirmer depuis de longues années. Il en est, d'ailleurs, une des meilleures incarnations dans tous les sens du terme ... Moi, je ne fais pas l'exégèse des propos du Président de la République-

s'exprimait- public composé du président du conseil régional, d'un président de conseil départemental et de parlementaires bretons -, a pris une position très nette.

laine. Vous souhaitez que nous modifiions la loi Littoral pour permettre de résoudre ce problème, qui, je vous l'accorde, est important pour l'environnement du Mont-Saint-Michel. Je ne pense pas que nous puissions intégrer cette belle construction intellectuelle dans le projet de loi. En revanche, je vous propose d'essayer de trouver des solutions concrètes et de voir avec les services de l'État

Ce qu'il vient de décrire est la réalité. À cet égard, monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir pris le soin de proposer une réflexion pour résoudre ce problème. Sachez

que le Mont-Saint-Michel attire chaque année 3 millions de visiteurs et que l'équilibre naturel de la baie nécessite la présence des moutons.

à M. Michel Vaspart. Cet amendement vise à clarifier le régime d'implantation de certains équipements d'intérêt public dans les communes littorales. Plusieurs situations de blocage sont connues, s'agissant, par exemple, des écoles de voile, des clubs nautiques ou des services d'assainissement. Aussi, un décret en Conseil d'État serait nécessaire pour fixer une liste des équipements nécessitant une proximité avec l'eau et le rivage, dont l'implantation pourrait s'effectuer

Cet amendement vise à exclure du champ d'application de la loi Littoral les équipements collectifs liés aux services d'assainissement, aux activités nautiques de manière large et à toute autre activité exigeant la proximité immédiate de l'eau, dont la liste serait fixée par décret. En l'état actuel du droit, certaines installations nécessaires à la sécurité publique, à la défense nationale, au fonctionnement des ports entre autres sont soustraites au principe d'aménagement de la loi Littoral lorsque leur implantation est dûment justifiée, en vertu de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, les stations d'épuration d'eaux usées non liées à une opération d'urbanisation nouvelle bénéficient d'un régime dérogatoire, conformément à l'article L. 121-5 du même code. outre, les constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques qui exigent la proximité immédiate de l'eau peuvent être implantées en dehors des espaces urbanisés de la loi Littoral, aux termes de l'article L. 121-17 du code précité.

pleinement justifiée. La délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou celle du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage et l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites garantissent le caractère équilibré de la dérogation. Il s'agit non

il sera rigoureusement impossible de faire quoi que ce soit sur ces

et les zones destinées à l'habitation qui prenne en compte la hauteur de l'éolienne, afin que la distance soit proportionnée à la taille de la structure. Le plan Climat fixe une ambition de neutralité carbone pour notre pays à l'horizon 2050 et de diversification des modes de production d'électricité. Le développement des énergies renouvelables, plus particulièrement de l'éolien terrestre, constitue un enjeu fort pour parvenir à cette évolution de notre mix énergétique et à la décarbonation de notre énergie. Ce développement doit toutefois être réalisé dans le respect des populations et de l'environnement. Pour que le développement de l'éolien ne s'accompagne pas de mise en danger de nos concitoyens, pour que le développement des parcs éoliens respecte l'acceptabilité des riverains, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il convient d'instaurer un éloignement proportionné

la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie de notre pays doit atteindre le seuil de 32 % en 2030. Si le développement du parc éolien participe à cet effort de diversification, il doit être encadré et doit respecter les paysages de nos territoires.

Pis, l'installation d'éoliennes à proximité immédiate de sites historiques met en péril la réalisation de certains projets de rénovation. La multiplication exponentielle et incontrôlée des projets éoliens inquiète clairement les élus locaux et la population.

en vue d'implanter le plus d'éoliennes possible sur leur territoire en raison des recettes fiscales induites, elles peuvent aujourd'hui regretter ces chantiers parfois hâtifs compte tenu des récriminations importantes des administrés, qui, non contents de devoir subir négativement l'effet visuel et sonore de ces structures au quotidien, doivent aussi faire face à la dévalorisation pécuniaire de leurs biens immobiliers. Alors que le législateur anglais et certains allemands ont opté pour une distance de 1 500 mètres et que certains États américains ont fixé une limite au-delà de 2 000 mètres mètres pour des raisons de santé publique, cet amendement vise à fixer une distance de 1 000 mètres entre les éoliennes et les habitations, ce qui permettrait de concentrer dans des zones inhabitées

Or je rappelle que l'éolien est une filière mature sur laquelle nous devons nous appuyer si nous voulons réussir la transition énergétique

rétablir une certaine sérénité dans l'hémicycle. Il ne s'agit pas du tout, monsieur Dantec, de contrecarrer l'extension des éoliennes.

il existe en France des personnes qui sont irrationnellement contre l'éolien. On les appelle d'ailleurs les anti-éoliens ! Avec tout le respect que je dois

éolicide. Je persiste également à rappeler que, en matière d'installation d'éoliennes, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment et n'importe où. La législation sert à encadrer, préciser et éviter les dérapages.

Il s'agit simplement de favoriser la revalorisation de ces sites, qui représentent des surfaces propices à l'installation de centrales photovoltaïques. Le territoire français compte en effet un nombre significatif de sites dégradés

ne peuvent aboutir, quand bien même ils auraient obtenu un avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ils sont en effet considérés comme une extension d'urbanisation en discontinuité de l'urbanisation existante.

les dispositions législatives actuelles permettent l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales en continuité des agglomérations et villages existants, à savoir des espaces comportant un nombre et une densité significative de constructions.

Cet amendement vise donc à adapter la loi Littoral, et plus particulièrement le régime des espaces proches du rivage, aux contraintes des activités agricoles de proximité, qui nécessitent uniquement la mise en place d'aménagements démontables et de faible importance.

pour des aménagements légers. Comme vous l'avez souligné, le SCOT, le schéma de mise en valeur de la mer, ou, en leur absence, l'accord du préfet après avis de la CDNPS,

autorise à déroger à la loi Littoral pour réaliser des constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement

les collègues ici présents qui représentent ces territoires pensent qu'il vaut mieux voter l'amendement du Gouvernement, je n'en ferai pas une affaire d'État, loin de là ! La parole est

concernant le traitement des déchets, de donner aux populations de ces quartiers et de ces villes une continuité en termes d'offre de service public, en particulier pour tout ce qui touche à l'environnement. Je suis favorable à ce que les agences des cinquante pas géométriques aient le plus de latitude possible pour pouvoir aménager, et qu'elles ne soient pas simplement cantonnées dans la remise de titres, tel que cela se passe aujourd'hui. Il existe un devoir d'aménagement ; dans le pays qui me concerne et que je connais le mieux, la Martinique, ces agences sont aujourd'hui

où s'applique la loi Littoral, une dérogation au principe d'extension de l'urbanisation au profit d'équipements d'intérêt collectif dont l'implantation est imposée par des nécessités techniques impératives, l'accord du préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. En effet, des contraintes d'ordre technique peuvent justifier que des équipements répondant à la satisfaction d'intérêts collectifs soient implantés en discontinuité de l'urbanisation existante, tout particulièrement dans les territoires ultramarins et insulaires, où la géographie est de nature à limiter les sites d'implantation potentiels de tels équipements. Ces contraintes techniques peuvent résulter de distances d'éloignement à respecter- c'est le cas -ou de la nécessité d'implanter un équipement, par exemple une station de potabilisation, à un endroit précis. En revanche, en l'absence de telles contraintes, une implantation en discontinuité, y compris pour des équipements d'intérêt collectif, est exclue. Cette dérogation ne saurait donc bénéficier à des équipements tels que des collèges, des installations sportives, etc., dont rien ne justifie qu'ils soient implantés à distance des zones urbanisées. Cette dérogation ne s'applique pas dans les espaces proches du rivage,

installation, et si nous estimons que la loi nationale n'est pas suffisamment adaptée à nos réalités, nous avons la possibilité de demander une habilitation.

En Corse, le secteur hôtelier génère 42 % des dépenses alors qu'il ne représente que 25 % de l'offre d'hébergement touristique et 40 % des emplois liés au tourisme. L'offre para-hôtelière, liée à la location non déclarée, notamment de résidences secondaires réalisées à cet effet, représente, selon les chiffres de l'INSEE, jusqu'à 75 % de l'offre en Corse. Cette réalité n'occasionne que peu de retombées sur le plan économique, et pratiquement aucune sur le plan social. Elle se traduit également par une hausse du prix du foncier et par une augmentation des défaillances dans le secteur : 75 établissements en 2017, soit une hausse de 70 % par rapport à 2010. Face à cette concurrence déloyale, seuls 20 % des établissements hôteliers de Corse disposent du nombre suffisant de chambres leur assurant une rentabilité pérenne. La moyenne insulaire est de vingt-neuf chambres, contre trente-six à l'échelon national, en raison de la faible implantation des chaînes hôtelières au profit d'établissements patrimoniaux.

égard aux dispositions adoptées en commission après l'article 12, il existe un risque important de remise en cause de la jurisprudence actuelle, qui octroie une possibilité d'extension limitée de l'offre hôtelière professionnelle existante. Cette disparition causerait un tort considérable à l'offre hôtelière professionnelle corse et à ses six cents établissements. Le présent amendement a donc pour objet de sécuriser juridiquement ces situations en transcrivant dans la loi la jurisprudence actuelle, c'est-à-dire en permettant l'extension limitée des établissements hôteliers, cette possibilité étant soumise aux prescriptions du PADDUC et à autorisation administrative, tout en évitant les effets d'aubaine en figeant les surfaces hôtelières à leurs emprises à la date de publication de la loi.

de réaliser des travaux d'extension dans la continuité de leur bâti, sans que ceux-ci ne puissent avoir pour effet d'accroître de plus de 50 % l'emprise foncière de ces établissements » ; 50 %, ce n'est quand même pas rien

biais de cet amendement, nous proposons d'exclure l'application du principe de continuité de la loi Littoral sur certaines zones caractéristiques du territoire montagnard

Nous nous sommes aussi engagés à veiller à la préservation de la philosophie de la loi Littoral et à n'envisager que des évolutions dûment justifiées et particulièrement encadrées.